concernés. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 1018, au sein de l’article 19.

les ventes et volumes de remboursement en France et à l’étranger. La plupart de ces informations sont couvertes par le secret des affaires et ne seraient pas utiles au CEPS dans la fixation du prix du médicament, dont je rappelle qu’elle dépend principalement de l’amélioration du service médical rendu, c’est à dire du progrès thérapeutique permis par le médicament. La majorité de ces informations ne seront pas davantage utiles au CEPS pour réguler les dépenses de médicaments. Lorsqu’elles sont utiles, elles lui sont d’ores et déjà transmises, par exemple pour documenter une demande de hausse de prix. Pour l’ensemble de ces raisons,

le montant de l’indemnité à verser par l’assurance maladie pour la distribution et la dispensation de spécialités du stock stratégique de l’État et des spécialités qui seraient achetées des achats conjoints européens.

Les travaux en cours dans le cadre de la révision du cadre législatif européen du médicament et les expériences passées montrent l’intérêt d’achats groupés au niveau européen pour des produits susceptibles de connaître

Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. Il permet également aux pharmaciens d’obtenir du laboratoire des informations sur la durée prévisionnelle des difficultés constatées. Cet amendement vise à consacrer l’existence de DP Ruptures dans le code de la santé publique, en clarifiant son pilotage et en complétant les missions du Cnop. La collaboration entre les pouvoirs publics et le Cnop prendra la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation.

par l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Ceux ci devraient, notamment, renseigner DP Ruptures sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Cela permettra de garantir une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaîne. En cas de non respect, des sanctions financières pourront être prononcées. à usage intérieur à une obligation de suivi des stocks qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, définira les conditions de cette obligation. Ces mesures contribuent à la mise en œuvre de l’une des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments,

Pour ce faire, il est proposé de ramener de deux ans à un an le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables.

L’on assiste depuis des années, et même depuis des décennies, à un gaspillage de médicaments, du fait notamment des soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels, comme les kits de pansements non utilisés. Le format des boîtes de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales et les kits de pansements qui excèdent les normes de 30 % à 70 % sont autant d’éléments qui expliquent cette situation. À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à accompagner la prescription de façon pragmatique. Tel est l’objet de cet amendement de mon collègue Daniel Chasseing.

des dispensations. Elle ne constitue pas non plus une solution appropriée face aux ruptures, puisqu’il n’est possible d’y avoir recours ni pour les formes injectables ni pour les formes pédiatriques, qui concentrent pourtant la majorité des risques de ruptures d’approvisionnement.

Mme Anne Souyris. Depuis la pandémie de covid 19, qui a nécessité de nombreuses dérogations ou adaptations à la législation sanitaire et sociale, certains médicaments mis à disposition en pharmacie de ville ou à l’hôpital font l’objet d’achats centralisés au niveau national, par Santé publique France, puis d’une mise à disposition gratuite aux pharmacies.

du Parlement sur les contrats d’achat liant l’État et l’industrie pharmaceutique.

n° 764 rectifié. Dans l’attente de la publication du décret désignant les CHU participant à l’expérimentation de retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, cet amendement vise à favoriser l’utilisation de dispositifs médicaux dont l’impact environnemental est susceptible de favoriser la transition écologique de notre modèle de santé et de réduire la pression sur les ressources limitées.

La commission soutient par exemple le déploiement de la remise en bon état d’usage. J’estime toutefois qu’agir sur le tarif de responsabilité des dispositifs médicaux n’est pas la bonne solution. L’assurance L’assurance maladie ayant avant tout pour objectif de solvabiliser les dépenses de santé les plus utiles pour les patients, il paraît en effet préférable que la base de remboursement par l’assurance maladie ne soit déterminée que par des facteurs d’ordre médical, à commencer par l’amélioration du service attendu, ou par des facteurs liés à la régulation économique. J’estime qu’il ne serait pas compréhensible qu’entre deux dispositifs médicaux similaires, le plus pertinent médicalement soit pris en charge sur une base plus faible

Cet amendement vise à obliger les entreprises à transmettre annuellement au CEPS, pour qu’il soit rendu public, le montant de l’ensemble des financements publics, directs ou indirects, et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Encore une fois, ces informations sont essentielles pour reprendre le contrôle sur nos produits de santé.

de produits selon l’utilisation que ces derniers en font. C’est d’autant plus inquiétant que, selon les documents budgétaires, « les services de l’assurance maladie ou un tiers de confiance désigné valideront la bonne adéquation

Souyris, pour présenter l’amendement n° 1121. Dès la première année des études de médecine, chaque étudiant apprend la fin du paradigme du paternalisme médical, les principes de la relation de confiance entre patient et soignant prescripteur, son impact sur l’utilisation du produit de santé soit ce qu’on appelle « l’observance » – et ses résultats sur la guérison du patient. Madame la ministre, dans cet article, vous opérez un retour en arrière. Désormais, la prise en charge d’un dispositif médical numérique sera soumise à à une justification de son usage par le patient. Cette logique d’infantilisation des patients nuit à la nécessaire relation de confiance entre le patient et son médecin. Ce dernier sera dans l’obligation de rapporter une utilisation considérée comme non pertinente à la sécurité sociale et d’arrêter la prescription du dispositif concerné. La transmission de ces données à un certain nombre d’acteurs, y compris aux fournisseurs de dispositifs médicaux, pose de nombreuses questions quant à la protection numérique du patient et au secret médical. Cette surveillance conjointe des patients et des médecins, dans la prescription, doit être remplacée par un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation des dispositifs par les patients, selon l’utilisation qu’ils en font et les besoins qui sont les leurs. Aucun calcul budgétaire ne doit justifier des mesures paternalistes et punitives telles que celles qui sont promues dans cet article. Nous appelons

que le prescripteur et le distributeur au détail soient informés sans délai de la suspension de la prise en charge du dispositif médical numérique par l’assurance maladie, afin de pouvoir réévaluer au plus vite la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre au bénéfice du patient.

reviendrait prioritairement aux professionnels de santé. Le prescripteur devra réévaluer la pertinence et l’efficacité de sa prescription, et pourra orienter le patient vers une offre d’éducation thérapeutique. Il s’agit de renforcer la capacité d’agir des personnes malades plutôt que d’aller trop précocement vers un abandon du dispositif médical pour celles – ce sont souvent les plus précaires – qui ont une faible littératie

cet amendement au nom de Corinne Bourcier. Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d’une surdité légère, qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde, qui empêche complètement la personne d’entendre la parole. Il n’existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité. Dans la prise en charge des surdités, le non usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé. En attendant que les pouvoirs publics épidémiologiques précises, cet amendement vise à inclure dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques la possibilité d’utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d’améliorer l’efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.

et de l’efficience des soins (Caqes). Elle recommande également une augmentation des moyens du CEPS pour réviser les nomenclatures des dispositifs médicaux, qui sont souvent obsolètes et source de dépenses inappropriées. Ce serait un bon moyen de diminuer les dépenses.

est ainsi libellé : La parole est à Mme la rapporteure. Cet amendement vise à conférer au dispositif de l’article 20 tout son caractère opérationnel en supprimant la phrase qui proscrit de faire varier le taux de participation de l’assuré à la prise en charge d’un dispositif médical en fonction des données d’utilisation. L’article 20 prévoit en effet de subordonner, dans certains cas, la prise en charge par l’assurance maladie à une utilisation effective du dispositif, ce qui suppose d’augmenter à 100 % le taux de participation de l’assuré. Quel est l’avis du Gouvernement ? Madame la rapporteure, vous souhaitez

santé solidaire ou de la protection universelle maladie. Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés faire remonter les données. Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante, alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous investissement chronique de l’État dans notre système de soins.

Ces modifications rendront opérationnelle cette remise en bon état d’usage, contribuant ainsi à l’économie circulaire – nous avons évoqué le sujet précédemment – et générant des économies pour l’assurance maladie.

dans le cadre d’une location, les dispositifs médicaux pouvaient, en réalité, déjà faire l’objet d’opérations de maintenance en vue d’une utilisation par un autre usager sans qu’il soit nécessaire de mobiliser le dispositif de RBEU. À titre d’exemple, la location des fauteuils roulants représente un montant

aux organismes d’évaluation de la conformité. Il s’agit alors bien de procédures de certification et non pas d’homologation, comme l’indique la loi à ce jour. Le terme « homologation » n’ayant pas de portée normative, il doit être modifié.

vise à intégrer dans les critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, plus spécifiquement quand celui ci est atteint d’une maladie chronique. En effet, la multiplication des dispositifs médicaux numériques incite à en différencier les apports pour les patients et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui, par définition, affecte durablement la vie quotidienne du patient. Près de onze millions de patients sont visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD, même si vingt millions de personnes, selon l’assurance maladie, ont recours à des soins liés à une pathologie chronique. Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de sa maladie par le patient. Pour ce dernier, il s’agit par exemple de

qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la sécurité sociale.

cet amendement est satisfait, puisqu’il est prévu réglementairement que la qualité de vie des patients soit intégrée par la HAS dans l’évaluation de l’intérêt

est à Mme Laure Darcos. Les dispositifs médicaux sont les seuls biens de santé non soumis à une franchise. En effet, les médicaments, les transports sanitaires et les actes médicaux, paramédicaux ou médico techniques sont tous soumis à ce mécanisme de participation de l’assuré. Cette exception n’est aujourd’hui justifiée ni par des arguments visant l’accès aux soins ni par des spécificités propres aux dispositifs médicaux, comme le démontre le rapport précédemment cité. En conséquence, cet amendement a pour objet de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d’un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuelle de 250 millions à 380 millions d’euros pour les comptes sociaux.

et même treize si l’on compte le geste exceptionnel de 150 millions d’euros qui avait été réalisé en 2024. Chacun de ces concours obéit à ses propres règles, dont certaines sont très datées, et l’ensemble ne permet désormais plus aucune lisibilité par rapport aux besoins des territoires ou de manière pluriannuelle. La présente mesure

plus de 80 % de l’enveloppe des concours de la CNSA. Nous pourrons ainsi mettre fin aux nombreuses procédures de remontée de données, qui embolisent les services départementaux, et et diriger tous nos efforts vers l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. En complément, l’enveloppe majorée des concours de la CNSA permet de garantir que les dépenses correspondant aux concours ainsi fusionnés seront compensées, pour chaque département, à hauteur strictement identique de celles de 2024. Nous tiendrons bien évidemment compte, pour ce qui est de l’APA, du geste exceptionnel de 150 millions d’euros autorisé par la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Je rappelle que ce dernier a permis à la quasi totalité des parents d’obtenir un taux de compensation de leurs dépenses d’APA d’au minimum – j’y insiste – 43 % en 2024. 2024. Un taux de compensation stabilisé sera ainsi garanti à chaque département en valeur relative, malgré une dynamique de dépenses qui n’a aucune raison de faiblir en 2025. Vous connaissez tous la problématique du vieillissement de la population et les prestations de compensation du handicap qui y sont associées.

Ce faisant, je le souligne, nous abandonnons des règles de répartition des concours entre départements, largement héritées d’une période antérieure à la création de la branche autonomie, qui avaient été établies à partir d’une enveloppe nationale indexée sur l’évolution des ressources de la CNSA. Dans le cadre de cette première étape de simplification, les concours

en avoir discuté avec le président du conseil départemental de La Réunion. Je suis tout à fait favorable à ce principe, mais je souhaiterais qu’il figure dans la loi. Certains territoires ultramarins, en effet, s’apprêtent à devenir les départements comprenant le plus de personnes âgées en France, alors qu’ils ont les taux de pauvreté les plus importants de France. Ces réalités structurelles impliquent donc une adaptation de certains paramètres des calculs de concours de la CNSA aux dépenses d’APA. Le sens de ce sous amendement est donc d’inscrire dans la loi que la majoration du taux de compensation selon un coefficient géographique bénéficiera aux outre mer. Quel

En conséquence, l’amendement vise également à adapter les modalités de l’évaluation du dispositif. Il prévoit qu’au plus tard, six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, réalisé avec l’appui de la CNSA, pour en dresser le bilan.

La frontière entre la prise en charge relevant des soins et celle au titre de la dépendance tend à s’effacer. L’amorce du virage domiciliaire et les progrès réalisés en matière de soutien à domicile permettent une entrée en en Ehpad beaucoup plus tardive. À l’heure où il est nécessaire d’assurer une prise en charge globale et continue, la distinction entre soins et accompagnement de l’autonomie apparaît donc artificielle.

entrait en contradiction avec les objectifs d’équité territoriale et de simplification propres à la branche. Ils appelaient donc, dès 2023, à une généralisation rapide de cette

Le montant des concours financiers de la CNSA leur étant attribué est minoré à ce titre. En conséquence, il est proposé d’adapter le calcul du montant des concours perçus par les départements expérimentateurs au titre de l’APA sur la durée de l’expérimentation. Ces modalités

L’article 21 décale la date butoir pour transmettre une candidature au 31 octobre. Or certaines informations nécessaires à l’instruction de cette décision ont parfois été communiquées tardivement. C’est le cas pour l’un des départements volontaires, qui n’a reçu ces informations que le 12 octobre. Il est donc souhaitable d’octroyer un délai supplémentaire.

l’amendement n° 509 rectifié. La Conférence nationale du handicap de 2023 prévoit la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale mise en place d’un nouveau parcours pour les enfants de moins de 6 ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant, de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neurodéveloppement.

Leur nombre, qui n’est pas connu avec exactitude, est estimé entre 6 000 et 8 000. La pénurie de médecins coordonnateurs tend à rendre encore plus incontournable le rôle de ces infirmiers en matière de coordination des soins et d’encadrement des équipes.

présent amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles, qu’il s’agisse des Ehpad, des crèches ou d’autres structures privées à but lucratif. Les dérives observées ces dernières années dans certains établissements sont alarmantes. De nombreux ouvrages et témoignages, notamment celui de Victor Castanet, ont mis en lumière des pratiques indignes : rationnement des repas, changement des couches espacé, maltraitance, etc. Des opérateurs privés à but lucratif intervenant auprès de publics vulnérables, nos aînés, nos enfants en bas âge ou encore des personnes en situation de handicap, se sont lancés dans une quête effrénée du profit au détriment de la qualité de la prise en charge. Face à ce constat, il est urgent d’agir. Si une réflexion plus globale doit être engagée sur la pertinence même de confier des pans entiers de nos politiques publiques à ces opérateurs, nous devons, dès à présent, fixer des limites. Cet amendement tend ainsi à conditionner l’attribution des financements publics à ces structures au respect d’une recherche raisonnable de bénéfices.

puisque vous ouvrez la possibilité de supprimer le financement des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, comment apprécier ce qu’est une « recherche raisonnable du bénéfice »

et à la Cour des comptes. Deuxièmement, la CNSA peut désormais procéder à la récupération d’indus jusqu’au niveau du groupe. Troisièmement, les contrôles peuvent s’appuyer sur la comptabilité analytique attestée par un commissaire aux comptes,

Sa mise en œuvre pourrait d’ailleurs s’avérer complexe, car des conventions collectives encadrent déjà les conditions de rémunération de certains cadres. Pour toutes ces raisons, j’émets également un avis défavorable.

l’heure, nous sommes bien conscients que, pour améliorer la situation de ces établissements sur le plus long terme, nous avons besoin de réformes structurelles.

plus de 50 % du financement des Ehpad ne dépend pas de la sécurité sociale, et c’est là où se trouvent les déficits. Je rappelle que les dotations des ARS ont augmenté de plus de 50 % depuis 2019, par comparaison. Sur ce sujet, et grâce au travail mené par les parlementaires avec l’appui du Gouvernement et compte tenu de la loi Bien Vieillir, nous allons déployer à partir du 1 janvier 2025 les tarifs différenciés dans un cadre national protecteur.

Elle permettra de faire converger vers le haut les financements consacrés à l’autonomie en Ehpad. Je remercie les vingt trois départements qui se sont portés candidats à l’expérimentation aux côtés de l’État, expérimentation dont nous venons de valider la réduction du délai à deux ans.

Houerou. Les prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) assurent des fonctions logistiques pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique, notamment à ses articles L. 6111 1 et suivants, qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé.

entre ces dernières et les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins. Quel

Les dispositifs et les prestations associées sont pris en charge par l’assurance maladie. En 2018, dernier chiffre connu, cela représentait près de 6,4 milliards d’euros. Il apparaît donc justifié de contrôler cette profession. Selon un rapport de l’Igas datant de 2020, il convient de renforcer les garanties en matière de qualité, de bonnes pratiques et de bon usage des ressources pour améliorer la confiance dans le secteur. une trop forte restriction des missions des PSDM ne me semble pas souhaitable, car ils assurent des prestations très utiles aux personnes, plus encore dans le contexte du virage domiciliaire. C’est donc un avis défavorable.

Nous sommes nombreux à nous faire le relais de nos territoires, élus, professionnels et citoyens, quand ils sont confrontés à des non sens administratifs, qui leur font souvent perdre du temps.

2017 – 2017 ! –, la députée Joëlle Huillier pointait déjà la nécessité de rendre le reste à charge du relayage soutenable, afin que tous les aidants puissent en bénéficier. Elle insistait ainsi sur le besoin de proposer un système financièrement acceptable.

sociale (CHRS) n’ont pas été revus à la hausse depuis quatre ans. Ces établissements – Ehpad, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales.

pour tout établissement d’hébergement pour personnes âgées, y compris privé à but lucratif, d’avoir un nombre minimal de places habilitées à l’ASH des personnes âgées.

95 % dans le public non hospitalier et 81 % dans le privé à but non lucratif. Dans le privé associatif, 91 % des établissements disposent de places habilitées, et trois Ehpad sur quatre sont habilités à l’aide sociale

concernant l’attribution des primes Ségur et Laforcade et des mesures salariales de la Conférence des métiers. En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous évaluation des besoins de financement de la prime Ségur. Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées sont durablement sous compensées par les financeurs du secteur, constituant l’une des premières causes du déficit desdites structures, avec l’inflation énergétique. Plusieurs financeurs ont d’ailleurs manifesté leur incapacité à compenser les organismes gestionnaires associatifs, faute de moyens octroyés par l’État. Face à cette situation très inquiétante pour l’équilibre financier de ces employeurs, nous estimons nécessaire que le Gouvernement dresse un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en chiffrant les sous financements de ces mesures salariales. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations. Cet amendement Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, l’une des organisations professionnelles représentant les employeurs de ces secteurs. Quel

11 milliards d’euros ! Elles bénéficient à un nombre très important de professionnels du secteur sanitaire et médico social. Ce montant a été calculé à partir de données statistiques robustes et intègre différents paramètres pour évaluer les compensations aussi précisément que possible, notamment les effets liés aux allégements généraux. Le versement par les ARS aux établissements a été réalisé sur la base de différents critères afin d’objectiver l’allocation des enveloppes.

Vous pouvez également vous rapporter aux éléments d’information sur les coûts des revalorisations qui figurent dans les annexes du PLFSS. Au regard de ces éléments, la remise d’un nouveau rapport ne me semble pas nécessaire. Avis défavorable.

est plus important dans le cadre de l’APA que dans celui de la PCH. Surtout, l’APA est une enveloppe fermée. C’est pourquoi, plutôt qu’une résolution au cas par cas, il est temps d’étudier la feuille de route et le coût pour une prestation unique au sein de la branche autonomie. Monsieur le ministre, je vous invite à lancer ce chantier.

La limite d’âge, en revanche, a été maintenue. Pour bénéficier de la PCH, il faut avoir eu une condition de handicap avant 60 ans, à l’exception des personnes qui exercent une activité professionnelle au delà de cet âge. L’APA présente des différences avec la PCH, notamment un plafonnement des plans d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie et une participation personnelle fixée en tenant compte des ressources du bénéficiaire.

Je l’ai dit devant vous à cette occasion, je ne peux que comprendre cette ambition de convergence face à de telles situations. Mais si l’on fait preuve de responsabilité, on ne peut que reconnaître qu’une suppression de l’APA au profit de la PCH pour tous

PCH a rappelé le débat théorique sur la légitimité même de la fusion des deux prestations. La situation est différente entre les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes dont l’ensemble du parcours de vie a été affecté par le handicap, y compris en matière de revenus. Pourrait on ainsi justifier l’absence de participation financière des personnes âgées restant à domicile, alors que leur situation patrimoniale et leur revenu n’ont, le plus souvent, rien à voir ? concertation Grand Âge et autonomie, remis par Dominique Libault en 2019, et le rapport de l’Igas de 2023 sur les défis de la politique domiciliaire n’ont ainsi pas remis en cause le principe de la distinction entre ces deux prestations.

au delà de laquelle il n’est pas possible de demander la PCH, y compris pour une cause apparue avant 60 ans. Pour ces raisons, il ne me semble pas pertinent de réaliser un nouveau rapport sur cette question. Je suis donc défavorable à votre amendement. Je mets aux voix l’amendement n° 806. L’amendement n°

de modernisation des Ehpad, notamment pour adapter ceux ci au défi de la transition écologique. La publication d’un rapport annuel sur les dépenses de l’Ondam allouées à la transition écologique serait un préalable utile. J’en viens à l’amendement n° 1287. En fonction de leur statut, les Ehpad acquittent des charges sociales et fiscales sur les salaires qui diffèrent.

et de cotisations sociales dans les Ehpad en fonction de leur statut. Il proposera des solutions pour mettre fin aux différences entre les régimes, au travers notamment de nouvelles modalités de financement. Quel

supplémentaires à destination des projets prêts à sortir de terre dans les Ehpad qui ont besoin de rénovation, dans une démarche d’isolation et de moindre consommation d’énergie. Enfin, pour aider les établissements à réduire leur empreinte carbone et à s’inscrire dans le dispositif Éco énergie tertiaire, nous finançons des postes de conseiller en transition

prévoit le versement anticipé de leur pension de retraite avec calcul sur les vingt cinq meilleures années. Cette méthode nous inquiète sur les induits et les trop perçus. Pourquoi ne respectez vous pas la loi que nous avons votée à l’unanimité,

une demande formulée par la profession agricole. Cet article procède à divers aménagements du code rural et de la pêche maritime qui permettent, à droit constant, d’unifier la présentation de ses dispositions législatives et de celles du code de la sécurité sociale.

et à expliciter certaines dispositions pour en faciliter la mise en œuvre par les caisses de sécurité sociale. Il est ainsi précisé que, pour les personnes ayant été affiliées au régime des personnes non salariées des professions agricoles à titre exclusif ou principal avant le 1 janvier 2016, les périodes d’assurance antérieures à cette date sont prises en compte, qu’elles soient cotisées ou assimilées. Il s’agit en outre de tirer les conséquences de la mise en place d’une assiette de cotisations unique, quel que soit le statut de non salarié agricole. à permettre la coordination légistique avec le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon. Enfin, il est proposé une adaptation terminologique dans la mention du dispositif de la pension d’orphelin.

propose d’étendre les nouvelles modalités de calcul de la durée maximale de cinq ans pendant laquelle une personne peut exercer une activité non salariée agricole en qualité de conjoint collaborateur aux personnes qui disposent de ce statut à compter du 1 janvier 2022 et jusqu’au 1 janvier 2025. Cette modification avait été votée par la commission des affaires sociales et jugée

; c’est pourquoi la commission des affaires sociales n’a pas pu se prononcer à son sujet. Cependant, il est identique à un amendement que nous avions voté en commission et qui avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40

le faire sous le statut de salarié. Cette requalification offre une protection sociale nécessaire à des aides familiaux qui se trouveraient, sans cela, dans une situation de travail dissimulé.

Il avait été prévu initialement que les pensions qui prendront effet entre le 1 janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seraient calculées de manière provisoire selon les modalités en vigueur

explications que j’estime nécessaires. Je me félicite que la réforme du mode de calcul de la retraite de base des non salariés agricoles, que nous attendons depuis de nombreuses années, aboutisse enfin.

qui représentent 85 % des non salariés agricoles, et 90 % des pensions liquidées. Les monopensionnés seront également gagnants. La pension de ceux qui ont les revenus les plus élevés était plafonnée par le barème de points de retraite proportionnel ; elle sera donc plus élevée qu’actuellement. à ceux qui ont des revenus plus faibles, et qui bénéficiaient pleinement de l’effet redistributif du barème de points, ils ne subiront pas de perte dans la mesure où leurs revenus seront rattrapés par la revalorisation de la pension majorée de référence sur le minimum contributif et servie par le régime général.

quelques détails techniques. Premièrement, la Mutualité sociale agricole (MSA) ne garde pas l’historique des revenus convertis en points antérieurement à 2016. Toutes les années cotisées avant 2016 seront donc liquidées sur les points, et non pas sur le revenu. Deuxièmement, il ressort des récents échanges que nous avons eus avec le Gouvernement et la MSA que les systèmes informatiques de liquidation des pensions devaient être révisés,

Le calcul de la pension de retraite basé sur les vingt cinq meilleures années de revenus ne sera possible qu’au terme d’une refonte du système informatique de la MSA, qui fonctionne actuellement en points. C’est pourquoi l’article 22 du présent PLFSS prévoit que les pensions liquidées entre janvier 2026 et le 31 décembre 2027 le seront selon le droit en vigueur

à revenir néanmoins sur la clause dite de sauvegarde, qui prévoit qu’à une date fixée par décret – au plus tard le 31 décembre 2028 –, les pensions feront l’objet d’un nouveau calcul afin d’être liquidées selon le droit réformé. Si le montant de la pension issue de ce nouveau calcul est supérieur à celui de la pension liquidée selon le droit antérieur, la différence sera restituée. Mais si la pension est plus faible, on ne recherchera pas le montant et l’indu ne sera pas réclamé. C’est bien clair.

Le Houerou. Notre groupe se réjouit également de la mise en œuvre de la réforme des retraites des non salariés agricoles au 1 janvier 2026

et de réversion des non salariés agricoles outre mer. Il s’agit d’une prolongation de l’habilitation inscrite à l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année dernière,

articles 3 et 5 . Au vu de la complexité de ce sujet et des potentiels impacts, non négligeables, pour les publics concernés, il convient que le Gouvernement présente des adaptations détaillées dans le corps de la loi et que les parlementaires puissent être consultés sur le sujet.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles dans l’Hexagone, et a permis au Gouvernement de de légiférer par voie d’ordonnance afin de rendre cette révision applicable aux exploitants agricoles ultramarins. L’application de cette réforme dans les territoires ultramarins est nécessaire

Néanmoins, nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique, alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer à se dégrader. Cet amendement vise donc à étudier la possibilité, sur la base du modèle existant pour le régime additionnel de la fonction publique, d’un nouveau modèle de financement des pensions pour les salariés et les indépendants, qui passerait par une capitalisation collective.

pour présenter l’amendement n° 319. Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire supporter la charge des efforts que l’État doit consentir par les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l’article 23 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en contradiction avec cette intention. en effet, en l’état, le report de la date d’indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non salariés agricoles. Cette mesure est problématique à plusieurs titres. En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l’État. L’indexation, sur une base régulière, des retraites sur l’évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur. En second lieu, cette mesure est d’une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50

une évolution sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d’inflation serait redevenu raisonnable. Les économies pour l’État, chiffrées à 3,6 milliards d’euros pour l’année 2025, proviennent donc d’une forme d’impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une simple variable d’ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires du passé. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 23.

à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quel que soit leur niveau de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. Cela s’appelle une baisse du pouvoir d’achat

et à multiplier les niches fiscales inéquitables. Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités percevant une pension modeste, qui sont souvent des femmes

rappelé, la situation très dégradée de nos finances publiques nous contraint à un effort ponctuel, qui sera partagé par l’ensemble de nos concitoyens. La participation des retraités à cet effort se traduit par une moindre revalorisation de leurs pensions de retraite que l’an passé, lorsque nous avions préservé les retraites du choc inflationniste en les revalorisant de 5,3 %. Tout le monde doit contribuer à hauteur de ses moyens, et les personnes qui touchent des pensions de retraite dont le montant est inférieur au Smic, soit 1 490 euros net,

des pensions – de base et complémentaires – n’excède pas le niveau du Smic sera ensuite revalorisé une seconde fois à hauteur de l’inflation constatée le 1 juillet 2025. Les retraités qui bénéficieront de cette seconde revalorisation percevront également en juillet un rattrapage du manque à gagner entre janvier et juillet.

Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires, aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables, notamment parmi les retraités. Pour cette raison, cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 100 euros brut et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites.